C'est le cas, notamment, du monde agricole, qui souffre actuellement d'une pénurie de main-d'oeuvre, le nombre de travailleurs saisonniers ayant fortement chuté en raison de l'épidémie. Pour faire face à cette situation, le Gouvernement a décidé d'allonger de six à neuf mois la durée pendant laquelle des travailleurs saisonniers étrangers peuvent exercer une activité professionnelle sur notre territoire, et ce à à titre dérogatoire, tant que l'état d'urgence sanitaire sera de mise. Nous aurions pu nous réjouir de cette mince avancée pour les travailleurs étrangers saisonniers, si celle-ci n'était pas due à une simple question conjoncturelle. Pour l'exécutif, le droit des personnes étrangères est uniquement une variable d'ajustement, n'ayant vocation à évoluer qu'en fonction des situations. Le Gouvernement ne fait que peu de cas de cette population migrante, simplement considérée comme de la main-d'oeuvre susceptible d'amortir les répercussions de la pandémie sur notre économie. Si des droits sont accordés, ils doivent être durables, et non conditionnés à l'urgence sanitaire. La rédaction de l'article 1 n'est donc pas satisfaisante, puisque le dispositif proposé ne revêt

par plusieurs autres États membres, de fixer la durée maximale annuelle de séjour en France des travailleurs saisonniers à six mois, pour s'assurer que leur résidence dans leur pays d'origine conserve bien sa qualité de résidence habituelle. L'extension à neuf mois doit rester ponctuelle, comme prévu dans la mesure qui vous est proposée. L'avis est donc défavorable.

en France au 16 mars -introduit une complexité inutile dans la gestion du droit au séjour. D'autres mesures que celles qui sont proposées par le Gouvernement ont été mises en place pour ces travailleurs, en particulier une simplification des démarches à effectuer pour bénéficier d'une autorisation provisoire de travail pour prolonger un contrat de travail ou en exécuter un nouveau. S'agissant de l'amendement n° 23,

Malheureusement, la pandémie liée au Covid-19 a rudement éprouvé notre économie. De nombreuses entreprises ont dû cesser leur production, faute d'activité. Comme tous les salariés en France, les travailleurs étrangers ont également été impactés. Or, pour ces populations, leur présence sur le sol français est conditionnée au maintien dans l'emploi. Sans activité professionnelle, il est à craindre que leur titre de séjour mention « travailleur temporaire » ne soit considéré comme caduc par les autorités françaises. Une telle situation serait injuste pour ces travailleurs dont la perte d'emploi ne serait due qu'aux circonstances sanitaires et non à un manque de compétences. Il est essentiel que, pour les travailleurs étrangers présents légalement sur notre territoire, la peur de l'expulsion et du chômage ne s'ajoute pas à l'anxiété engendrée par la pandémie. Ainsi, il est proposé à travers cet amendement que la perte d'un emploi en raison de l'épidémie de Covid-19 ne puisse être opposée au renouvellement du titre de séjour des travailleurs temporaires pendant l'état d'urgence sanitaire, et dans un délai de six mois à compter de la fin de celui-ci. Une telle proposition devrait permettre de sécuriser la situation des salariés étrangers présents actuellement en France.

Par ailleurs, cet amendement aboutit à une prescription formulée de manière trop générale et dont les contours sont insuffisamment précis, ce qui donnerait lieu et matière à de nombreux contentieux. Dans le contexte de l'épidémie, et compte tenu de ses effets sur l'économie, il est évidemment attendu de l'administration, dans le cadre de l'examen de l'ensemble de la situation

en permettant un droit de tirage, si je puis dire, sur les caisses de retraite des indépendants pour financer des aides sociales. Certes, monsieur le rapporteur

la validation législative des décisions prises par les instances décisionnelles des régimes de retraite des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux, alors que ce sont ces instances elles-mêmes qui ont souhaité apporter un soutien à leurs assurés en difficulté. Monsieur le rapporteur pour avis, vous dites que nous avons été mis devant le fait accompli, mais, après tout, ces instances ont délibéré librement,

est meilleur ! Nous proposons une nouvelle rédaction de l'article 1 AA, afin de mieux préciser les conditions de mobilisation éventuelle des réserves des régimes complémentaires des indépendants en inscrivant dans la loi clairement des critères de soutenabilité à préserver pour ces derniers. Ceux-ci concernent ainsi le niveau des réserves à l'issue du prélèvement éventuel, la liquidité des actifs permettant d'assurer les échéances de prestations ou encore les conditions de cession des actifs.

Vous justifiez le maintien de ce dispositif et son encadrement par le fait que des caisses de retraite s'y sont déjà engagées.

de l'ensemble de ces caisses ont un objectif : assurer les retraites de celles et de ceux qui ont cotisé. En dérogeant à cette règle, comme le disait notre collègue Monique Lubin, vous enfoncez un coin, vous créez un précédent, et rien ne nous garantit

Ce ne serait pas la première fois que vous contesteriez une décision prise par des partenaires sociaux. Si vous considérez que c'est une erreur, monsieur le ministre, il faut l'assumer et revenir dessus.

La rédaction adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale permet de créer de manière permanente des droits au profit des salariés, et non pas seulement pour la période de crise sanitaire. La pérennisation de la validation des droits à la retraite au titre de au titre de l'activité partielle indemnisée se justifie d'abord pour des raisons d'équité. En effet, les périodes de chômage sont réputées assimilées dans la prise en compte des trimestres de retraite. En outre, le recours à l'activité partielle, certes massif en ce contexte de crise sanitaire- nous en avons parlé longuement longuement cet après-midi -, n'est pas seulement un dispositif de crise ; des ruptures de droits peuvent survenir- cela a déjà pu être le cas dans quelques situations plus marginales, mais réelles. Un dispositif pérenne sera plus protecteur pour les salariés. Enfin, en tout état de cause, le coût de cette mesure financée par le FSV devrait être limité. La parole est à M.

Dans sa rédaction initiale, l'article 1 A visait à sécuriser les droits sociaux des travailleurs dont l'activité est partielle, en permettant de créer, de manière pérenne, des droits à la retraite au titre des périodes correspondantes. Il s'agissait d'un dispositif particulièrement bienvenu. Or la commission l'a restreint aux périodes d'activité partielle comprises entre le 1mars 2020 et le 31 décembre 2020, non sans risque pour la prise en compte des difficultés de certains secteurs comme l'agriculture ou la restauration, qui, nous le savons, se prolongeront probablement au-delà de la seule année civile 2020. Cet amendement a donc pour objet de rétablir l'article 1 A dans sa rédaction initiale, en supprimant cette limitation dans le temps.

complémentaire mise en place dans les entreprises au profit des salariés et permettre de reporter le paiement des primes et cotisations correspondantes. Des conventions collectives et des contrats d'assurance prévoient que les garanties des salariés sont suspendues dans le cas où leur contrat de travail Dans le contexte du recours massif à l'activité partielle, qui emporte la suspension du contrat de travail, cette situation n'est pas acceptable. Le Gouvernement entend garantir que les salariés resteront bénéficiaires notamment de leur couverture santé ou prévoyance mise en place dans l'entreprise. Ainsi, cet amendement tend à rendre obligatoire, depuis le 12 mars et jusqu'au 31 décembre 2020, le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés en activité partielle, indépendamment des conventions, accords et décisions unilatérales de l'employeur, ainsi que des clauses des contrats d'assurance. Le non-respect de ces dispositions législatives dérogatoires aurait pour conséquence de priver le régime d'entreprise mis en place du bénéfice des exemptions de cotisations sociales liées à la mise en place des garanties. L'amendement prévoit des dispositions d'ordre public par défaut pour les régimes dont les cotisations et les prestations sont assises sur la rémunération soumise à cotisations sociales. L'indemnité d'activité partielle brute mensuelle constituera l'assiette minimale pour le calcul des primes ou cotisations d'assurance, ainsi que des prestations. Les employeurs seront ensuite libres de proposer une assiette plus importante et de proposer une répartition entre les salariés et les employeurs plus favorable aux salariés. Enfin, l'amendement tend à permettre aux salariés et aux employeurs de bénéficier jusqu'au 15 juillet prochain, sans frais ni pénalités, de reports et de délais de paiement des primes et cotisations dues depuis le 12 mars auprès de l'organisme assureur, avec interdiction pendant cette période de résilier les contrats d'assurance et de suspendre les garanties en cas de défaut de paiement des primes et cotisations. Les employeurs et salariés devront ensuite s'acquitter des paiements suspendus ou reportés dans la limite de deux échéances simultanées, sous réserve que l'ensemble des échéances aient été honorées au 31 décembre 2020. Quel est l'avis de la commission des affaires

partout dans le monde. Plus de 3 millions de Français, vous le savez, sont établis hors de France. Une des premières mesures qui avait été adoptée lors du premier texte relatif à l'état d'urgence sanitaire avait été

Monsieur le ministre,

le cumul intégral et lève le critère de carence applicable. Une instruction similaire a été donnée à la CNRACL par le Gouvernement. Si le Gouvernement partage le souci de la commission de régulariser juridiquement le dispositif mis en place, il conviendrait qu'il soit rédigé en termes plus généraux

plutôt poser une question. À titre personnel, je suis favorable au cumul emploi-retraite pour les personnels soignants

Cet article permet aux étrangers séjournant en France dont les documents de séjour arrivent à échéance entre le 16 mai et le 15 juin 2020 de les prolonger de 180 jours, soit six mois. Certains étrangers qui, pour des raisons prévues par notre droit commun déjà bien laxiste, voyaient leurs documents de séjour arriver à expiration le 15 juin auront le droit d'être sur notre territoire jusqu'au 15 décembre. Quel est le rapport entre le mois de décembre et la fin de l'état d'urgence début juillet ? On se le demande ! De plus, l'article L. 311-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit déjà une dérogation de trois mois après expiration dans certains cas et pour les étrangers ayant un titre de séjour pluriannuel. Cette disposition vise donc la filière préférée des mondialistes : celle des demandeurs d'asile, qu'on ne déboute jamais vraiment de ce droit tout en le galvaudant. Cette tendance est consternante : toujours plus de laxisme, jamais plus de fermeté ! Vous auriez pu proposer, par exemple, de faire respecter le droit français et d'expulser au moins les déboutés testés positifs au Covid-19. Les frontières ne sont pas une aberration sanitaire. Cette affirmation assénée sans explication est contraire au bon sens élémentaire et démontre l'entêtement idéologique de nos dirigeants. Pourtant, c'est bien entre les quatre murs de nos appartements qu'ils ont décidé de nous confiner, érigeant de nouvelles frontières à nos libertés sans que nous le contestions. Cela s'appelle être pragmatique ! Nous aurions peut-être pu éviter cette crise ou en limiter les effets si nous avions appliqué le principe de précaution de protection aux frontières. Pour des raisons sanitaires et sécuritaires évidentes, le contrôle de l'immigration doit être effectué dans le cadre strict prévu par la loi. La situation d'urgence actuelle ne justifie pas de succomber à la facilité administrative en prolongeant la validité des documents de séjour pour une durée de six mois.

et qui sont dans l'incapacité d'en demander le renouvellement du fait de l'arrêt du fonctionnement des préfectures. Eh oui ! Afin que ces personnes en situation régulière ne se retrouvent pas en situation irrégulière

Le présent article prolonge les différents types de titres de séjour dont bénéficient les personnes étrangères pouvant ou ayant pu expirer entre le 16 mai et le 15 juin 2020. Ainsi est prolongée pour 180 jours la validité des visas de long séjour, des titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger, des autorisations provisoires de séjour et des récépissés de demandes de titres de séjour. Les attestations de demande d'asile bénéficieront, elles, d'une prolongation de leur validité pendant 90 jours. Nous saluons ces décisions, qui semblent aller dans le bon sens. Deux éléments nous interpellent cependant. Tout d'abord, nous ne jugeons pas nécessaire de marquer une différence entre les attestations de demande d'asile et les autres types de séjours en termes de durée de leur validité. Le présent amendement vise par conséquent à harmoniser cet élément afin que tous les titres et attestations de séjour bénéficient d'un renouvellement de leur effectivité pour 180 jours. il est à craindre que la date du 15 juin ne soit précipitée. Les préfectures sont surchargées de demandes multiples ; elles pourraient ainsi ne pas avoir repris une activité normale à cette date. Par prudence, nous proposons de repousser cette échéance au 10 juillet, soit à la fin prévue de l'état d'urgence sanitaire, prolongé par la loi du 11 mai 2020. Cette disposition devrait permettre aux préfectures de gérer au mieux leur charge de travail et de ne pas traiter les demandes des étrangers dans une hâte contre-productive. L'amendement

Depuis le 11 mai, les Français ont retrouvé une relative liberté. Il est pour l'heure difficile d'évaluer l'impact de cet événement sur la circulation du coronavirus parmi nos concitoyennes et nos concitoyens. Le risque d'une deuxième vague n'est pas à négliger, de nouveaux semblant en effet se déclarer dans des abattoirs et des écoles au sein de zones pourtant classées vertes. À la lumière de ces éléments, un nouveau pic de la pandémie est à craindre, même si nous espérons que ce ne sera pas le cas. Une telle éventualité signifierait probablement le reconfinement de la population au mois de juin et pour une durée indéterminée. Cela engendrerait une incapacité de nos préfectures à traiter les demandes des personnes migrantes dans des conditions adéquates. Afin de permettre la décongestion progressive des services préfectoraux, il est proposé par cet amendement de décaler la date d'expiration des titres de séjour du 15 juin au 4 septembre. Une telle proposition permettrait de sécuriser les droits des étrangers susceptibles de se trouver en situation irrégulière au cours de l'été tout en donnant aux préfectures la possibilité

alors nous dire : j'avais raison ! Je propose dans l'immédiat, s'agissant d'une dérogation, qu'elle soit strictement limitée en raison des éléments qui nous sont donnés, c'est-à-dire un redémarrage au 15 juin avec un surcroît de personnel. J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble des amendements.

de proroger ou de prolonger la durée de validité des titres arrivant à expiration entre le 16 mai et le 10 juillet, ou le 4 septembre. Le Gouvernement ne souhaite pas que cette prolongation soit différente en ce qu'elle prolongerait les attestations de demande d'asile de 180 jours et non de 90 jours.

ou un permis de séjour temporaire aux titulaires d'un visa de court séjour et aux personnes exemptées de visa qui sont obligés de rester au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Quel est l'avis de la commission ? Ces deux amendements

Tout au long du confinement, des associations comme la Cimade n'ont eu de cesse de nous alerter sur la précarité grandissante des personnes migrantes, notamment les plus jeunes entrés dans l'âge adulte depuis peu. semblent être les plus démunis, parce qu'ils ne sont souvent pas accompagnés de leurs parents. Ils n'ont, par ailleurs, pas acquis une expérience de vie solide qui leur permettrait de mener bien leurs démarches administratives. Autonomes par le droit, en raison de leur âge, ces jeunes adultes migrants ne le sont pas dans les faits. Le présent amendement a pour objet de leur offrir une relative stabilité en délivrant automatiquement une autorisation provisoire de séjour aux personnes accédant à la majorité. Il est également proposé de fournir un récépissé de demande de titre de séjour à ceux qui atteignent l'âge de 19 ans pendant l'état d'urgence sanitaire. Il n'est pas acceptable qu'à la peur de l'expulsion s'ajoute celle engendrée par l'épidémie de coronavirus. Une telle mesure devrait donc permettre aux jeunes migrants d'aborder avec moins d'inquiétude leur séjour sur le territoire français. Quel

Les dispositions introduites supprimaient toute référence législative au récépissé dans le Ceseda, au profit d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour. Cette suppression est issue d'une volonté de déployer un nouveau service de dépôt en ligne et d'instruction dématérialisée des demandes de titres de séjour. Ce procédé pose trois problèmes majeurs. Tout d'abord, le déploiement de la dématérialisation pénalise les étrangers. Exposées à une grande précarité, ces personnes ont souvent des difficultés pour accéder à internet. Afin de ne pas rompre l'égalité entre les requérants étrangers, il est impératif de maintenir un caractère facultatif aux procédures en ligne. Ensuite, la rédaction de l'article proposée par M. Buffet renvoie au domaine réglementaire la délivrance des récépissés. Alors que nous nous battons aujourd'hui pour éviter que l'exécutif n'ait systématiquement recours aux ordonnances, il est paradoxal que le Sénat souhaite se dessaisir d'un domaine législatif qui lui revient de droit. Enfin, le Ceseda prévoit qu'un récépissé autorise légalement les personnes à séjourner sur notre sol, mais aussi et surtout à voyager, à travailler ou à accéder à des avantages sociaux. Lui substituer un simple document provisoire aux contours flous ne garantit aucunement qu'il n'y aura pas, en l'occurrence, d'atteinte aux droits des étrangers. En l'état, nous ne pouvons soutenir cet article. Je suis saisie

de séjourner en France sans attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, et sans récépissé clairement établi, mais simplement avec un document provisoire qui leur permettrait, par ailleurs, d'exercer une activité professionnelle. Je vous trouve bien timorés finalement, mes chers collègues. Tant qu'on y est, abrogeons tout papier d'identité ! Comme cela, tout le monde pourra venir dans notre beau pays ... Vous serez enfin heureux

Cette violence, n'en déplaise à une artiste sans talent et sans public, ... Ouh ! ... n'est pas le fait de la police, dont je salue le travail, mais de la racaille qui y vit et qui déteste tout ce qui peut incarner la France. Nos compatriotes continueront, eux, de se pousser pour faire de la place aux autres, et vous vous féliciterez de toute cette diversité que vous ne voyez qu'à la télé ou dans les bureaux de vote, clientèle bien fidèle et pour l'instant docile. La facilité administrative et les aménagements dérogatoires vis-à-vis des étrangers menacent d'aggraver la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons. L'urgence impose la prudence en matière sanitaire et sécuritaire, ce qui implique des règles claires et un cadre strict. De plus, la possibilité d'exercer une activité professionnelle avec un simple document provisoire peut accentuer le phénomène de création de faux documents. De telles mesures risquent d'entraîner une confusion administrative au niveau des entreprises et du suivi par l'État. On nous avait promis des changements après cette crise sanitaire, les voici : toujours plus de laxisme pour les filières d'immigration et un déséquilibre démographique encouragé ! Le confinement n'est toujours pas terminé pour nos restaurants, bars et cafés, ces lieux de vie qui sont au coeur de nos modes de vie. Encadrés par les contraintes, surveillés et contrôlés de près, tous ces petits patrons devront faire des efforts surhumains pour relancer leur activité. Dans le même temps, M. Castaner continue à accueillir toute la misère du monde et Mme Belloubet ouvre les centres de détention. À l'image de cette France qui se retrousse les manches, envers et contre tout, je ne me résigne pas : je demande la suppression de cet article ajouté par la commission des lois à majorité, rappelons-le, Les Républicains.

de renvoyer au pouvoir réglementaire, dont elles relèvent, les modalités de délivrance par l'administration d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de titre de séjour ou lors de son renouvellement. Il s'agit donc

En deuxième lieu, la dématérialisation des procédures administratives pose un grand nombre de problèmes à beaucoup de publics, et on peut imaginer assez aisément que les personnes concernées par les demandes de titre de séjour ne sont pas parmi celles qui accèdent le plus facilement à l'outil numérique.

il n'est pas nécessaire d'ajouter des difficultés aux personnes concernées. En troisième lieu, enfin, il me semble que le récépissé de demande de titre de séjour n'est pas seulement cité dans la partie législative du Ceseda, il

pour demandeur d'asile (ADA) pour les personnes étrangères qui auraient cessé d'y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Nous ne pouvons que saluer une telle décision, l'ADA permettant à plusieurs milliers de personnes migrantes de recevoir quotidiennement un revenu. Cette somme est souvent la seule qui leur est attribuée et qui leur permet de survivre. Cet article nous donne par ailleurs l'occasion d'appeler l'attention du Gouvernement sur un problème qui pourrait bientôt se poser aux étrangers bénéficiaires de cette allocation. En raison de l'obsolescence programmée des cartes de paiement de l'ADA, l'Office français de l'immigration et de l'intégration devra remplacer 60 000 de ces cartes d'ici à la fin du mois d'août. Afin de pouvoir récupérer leur moyen de paiement, les personnes bénéficiant de l'ADA seront donc convoquées prochainement par les directions territoriales de l'OFII. dans certaines régions particulièrement vastes, comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine, les directions territoriales sont peu nombreuses.

nous espérons que le Gouvernement mettra en place un régime dérogatoire, afin de permettre aux demandeurs d'asile de bénéficier de leurs droits, tout en respectant les préconisations gouvernementales en matière de trajet autorisé. L'amendement

La maîtrise des dépenses coûteuses, et même ruineuses quand il s'agit de l'immigration, est une nécessité impérieuse. Les mesures dérogatoires en matière de droit d'asile ne font qu'alourdir le coût de la crise et aggraver ses conséquences économiques et sociales.

étude du CEPII, service de recherches économiques rattaché au Premier ministre, Édouard Philippe, publiée en 2018, a estimé le coût de l'immigration à 1,65 point du PIB annuel sur trente ans, ce qui représente 40 milliards d'euros par an. Et encore, l'étude en question s'arrête en 2011 ; cela fait donc sûrement beaucoup plus Au moment où la Commission annonce une chute de 8,2 % de notre PIB, je crois que nous avons trouvé une belle source d'économie structurelle pour éviter la crise, sur le court et le long terme. Cette solution exige des frontières et de l'ordre, mais, pour cela, il faudrait au moins une crise sanitaire grave et deux mois pleins de confinement pour vous retirer vos oeillères idéologiques. Tout cela a bien eu lieu, mais rien n'y a fait ; l'autre, toujours l'autre, avant les nôtres ... Malgré tout, je vous demande, mes chers collègues, de montrer que le bon sens reprend ses droits dans cet hémicycle, en votant cet amendement. Quel est l'avis de

si vous voulez faire preuve de pragmatisme, vous rejetterez l'amendement qui vient de vous être présenté. Cela dit, je ne vous demande même pas de faire preuve de pragmatisme ; je vous demande, tout simplement, de faire preuve d'humanité, en ne laissant pas en France, sur notre territoire, des gens

simplement rappeler que les bénéficiaires de l'allocation pour demandeur d'asile, une allocation de subsistance versée sous conditions de ressources, font manifestement partie des personnes en situation de pauvreté bénéficiaires des prestations sociales durant la période d'état d'urgence pour lutter efficacement contre la propagation du virus sans dégrader les conditions de vie des personnes précaires. Les demandeurs d'asile qui auraient dû quitter le lieu d'hébergement mis à leur disposition ont été exceptionnellement autorisés à s'y maintenir, par cohérence avec ces mesures d'accompagnement. Il est nécessaire d'éviter toute rupture du versement de l'ADA, qui constitue, pour ces personnes, l'unique source de revenus, l'unique moyen de subsistance. En outre, la mesure est proportionnée

vous ne nous avez pas convaincus. Une fois que j'ai dit cela, j'ai une question à vous poser, monsieur Ravier. Puisque les étrangers sont votre fonds de commerce, vous êtes-vous

pour mettre en place un dispositif d'intéressement, par une décision unilatérale de l'employeur. Nous nous étions déjà opposés à cette disposition, de notre position, nous demandons la suppression d'un dispositif qui vise à justifier l'absence de revalorisation des salaires par l'association au résultat de travailleurs et de travailleuses qui ne sont pas décisionnels dans les orientations de l'entreprise. De plus, ce dispositif est extrêmement coûteux pour la sécurité sociale,

ou même l'application d'un contrat d'intéressement, ne semble pas justifié. Faisons le calcul : la durée d'un contrat d'intéressement étant de trois ans, cela reviendrait à priver de ce dispositif les entreprises ayant conclu un contrat d'intéressement au cours des huit dernières années,

Il est en effet particulièrement difficile à ces entreprises de négocier des accords d'intéressement. L'amendement n° 234 rectifié vise, d'une part, à élargir aux entreprises de

La commission estime que la dérogation au principe de la mise en oeuvre de l'intéressement par accord n'est justifiée que pour les très petites entreprises.

et de réduire de cinq à deux ans la période entre la dernière conclusion d'un accord et la date d'effet de mise en place, par décision unilatérale, d'un nouvel intéressement. L'intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale, qui fait l'objet d'une négociation collective par les partenaires sociaux,

dernière possibilité ne permet pas d'avoir une couverture suffisante des entreprises concernées. C'est d'ailleurs pour cela que la mesure avait été initialement proposée. En effet, seulement 3,2 % des salariés des entreprises de un à neuf salariés étaient couverts par un accord d'intéressement en 2017, contre plus de 10 % dans les entreprises de dix à quarante-neuf salariés et environ 70 % dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. Bien que le taux de couverture de l'intéressement demeure relativement faible dans les entreprises de dix à

au travers de l'article 1 . Par ailleurs, il convient de noter que, pour inciter les PME de onze à cinquante salariés à mettre en place l'intéressement, des mesures ont été prévues par la loi Pacte, notamment la mise en place d'accords types par branche professionnelle, auxquels elles peuvent adhérer par décision unilatérale. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par des accords de branche, des accords types d'intéressement ont également été créés par le Gouvernement, afin de faciliter la négociation et la conclusion des accords. La mesure doit également être limitée à la mise en place de l'intéressement pour la première fois,

En outre, les entreprises qui ne rempliront pas la condition de délai de cinq ans auront toujours la possibilité de conclure un accord selon les modalités de droit commun. Elles ne seront donc pas privées de l'accès à l'intéressement. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

peut bénéficier d'un avis favorable du Gouvernement. La possibilité de mettre en place un régime d'intéressement par décision unilatérale est une mesure d'amorçage et doit donc être limitée à la mise en place de l'intéressement pour la première fois. Le Gouvernement a également émis un avis défavorable

Or comment faire lorsque l'on n'est pas certain de son résultat en fin d'année, parce que l'on est quand même dans une période de perturbation économique ? La mise en place de l'outil de l'intéressement, dans ce contexte particulier, est un bon outil. En revanche, il nécessite un aménagement lié à la crise ; c'est l'esprit même de l'amendement proposé. Je soutiens donc complètement vos arguments,

Par conséquent, dans le régime de l'intéressement, des conditions particulières pouvant justifier cette dérogation à la distribution de revenus aux salariés

hypothéquer les possibles hausses de salaires à venir, mais nous entendons tout de même permettre ici et maintenant aux salariés de notre pays qui n'ont pas la chance de bénéficier d'un accord d'entreprise d'avoir accès à l'intéressement.

sur la voie d'une prise en compte de cette aspiration de nos concitoyens à plus de revenus, aspiration qui s'est également manifestée par une demande très forte à pouvoir bénéficier d'heures supplémentaires exonérées de charges sociales et fiscales. Il est